Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation ?

M. le ministre de l'éducation nationale. Lors du précédent quinquennat a été mis en place, à partir de 2014, un dispositif inédit : les conventions pour une politique en faveur de l'école rurale et de montagne. Le 24 janvier de cette même année, le Cantal était le premier département à signer ce type de convention. Promouvant une approche de concertation nouvelle, ces conventions prévoient l'accompagnement des territoires ruraux fragilisés par la baisse démographique en préservant l'existant et en apportant des moyens supplémentaires en personnels enseignants, au profit des collectivités. De leur côté, les élus s'engagent à conduire au niveau local une réflexion sur le réaménagement des réseaux d'écoles. s'agissait de construire une école rurale de qualité et de proximité, qui s'émancipe de la menace récurrente des effets comptables résultant de la démographie. Deuxièmement, il s'agissait de maintenir un climat de travail serein et constructif entre les élus et les autorités académiques, au profit de la communauté éducative locale.

L'État a accompagné cette démarche en apportant de la visibilité, des conventions triennales renouvelables, et en limitant le nombre de suppressions d'emploi, puisque pour la première fois, sur deux cartes scolaires consécutives, des dotations « ruralité » avaient été fléchées. Alors que, pour les premières de ces conventions, signées en 2013-2014, approche l'échéance du renouvellement, et tandis que des départements qui avaient souhaité se donner un temps de réflexion envisagent à présent de s'engager dans la démarche, je souhaiterais, monsieur le ministre de l'éducation nationale, connaître les dispositions que vous comptez prendre

Au-delà des conséquences économiques et sociales auxquelles cette mobilisation générale a tenté d'apporter des réponses, il a été admis que cet épisode de gel a montré l'absolue nécessité d'un développement de la couverture assurantielle pour les viticulteurs. Devant la multiplication des aléas climatiques, les viticulteurs, mais également tous les autres agriculteurs, doivent intégrer la gestion des risques dans la conduite de leur exploitation : le gel et la grêle sont des risques assurables non négligeables être intégrés de façon prioritaire dans la réflexion économique sur le développement des entreprises viticoles. Si les systèmes d'assurance proposés ne correspondent pas forcément aux attentes des viticulteurs, en particulier à celles des propriétaires de petites exploitations, ils restent le meilleur rempart face à une telle catastrophe économique. seuls 20 % des viticulteurs sont assurés et peuvent le faire : cette très faible proportion traduit les imperfections, les insuffisances et, surtout, le coût exorbitant du système assurantiel actuel. Les tarifs très élevés, conjugués à un taux de franchise de 25 %, n'autorisent pas les petits propriétaires à se protéger contre les risques. Comme le souligne Bernard Artigue, président de la chambre d'agriculture de la Gironde, « il est primordial de remettre sur la table tous les éléments pour améliorer le système d'assurance d'ici à la prochaine campagne et de le rendre plus attractif Monsieur le ministre, je me dois d'être le porte-parole à cette tribune de trop nombreux viticulteurs de la Gironde qui doivent faire face à une situation préoccupante en multipliant les efforts pour maintenir l'activité de leur exploitation et contribuer ainsi à la survie de nos territoires ruraux. Vous reconnaîtrez que, pour ces viticulteurs, les tarifs prohibitifs de l'assurance représentent un frein à la souscription. Seule la solidarité nationale est en mesure de redonner espoir à toute une profession ! À la suite de cet épisode catastrophique, quelle réponse pensez-vous pouvoir apporter à ces viticulteurs en grande souffrance ?

a connu deux épisodes de gel qui ont affecté un grand nombre de régions et différents types de productions. Plusieurs dispositifs peuvent déjà être mobilisés dans les différentes filières : recours à l'activité partielle pour les salariés, dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti si les pertes sont avérées, demande de report du paiement des cotisations sociales auprès des caisses. Par ailleurs, afin de prendre en compte le caractère spécifique de la viticulture, le dispositif de prise en charge partielle par l'État à hauteur d'un tiers des frais de restructuration des prêts professionnels vient d'être élargi aux viticulteurs et prolongé jusqu'au 31 décembre 2017. Les viticulteurs ont également accès au dispositif de prise en charge du coût de la garantie bancaire octroyée pour les prêts de restructuration de l'endettement bancaire ou de renforcement du fonds de roulement, qui est également prolongé jusqu'au 31 décembre 2017. Si les pertes de récolte ne sont pas éligibles au régime d'indemnisation des calamités agricoles, les pertes de fonds consécutives à une taille sévère à la mortalité des jeunes ceps peuvent malgré tout être indemnisées. Les préfets réuniront prochainement les comités départementaux d'expertise pour que ces derniers rendent leur avis sur le caractère de calamité agricole des Si le caractère exceptionnel des variations de température est confirmé, je reconnaîtrai rapidement le caractère de calamité agricole. En outre, des mesures de gestion de crise complémentaires destinées au secteur viticole sont également développées pour conforter la résilience des exploitations. Il en est ainsi de la possibilité, pour pour les viticulteurs affectés par des sinistres climatiques, d'acheter dans certaines conditions des vendanges à d'autres producteurs afin de compléter leur récolte. Sur le plan plus général de l'équilibre des marchés, le secteur viticole et celui des spiritueux sont de formidables moteurs pour faire rentrer des devises dans l'économie française. L'un et l'autre assurent une part très importante de l'excédent commercial français. L'état des lieux de notre agriculture qui a été dressé jeudi 20 juillet, lors du lancement des états généraux de l'alimentation, l'a démontré. Il faut néanmoins souligner que les importations françaises de vin sont en augmentation. C'est notamment le cas pour les vins espagnols, et cela déstabilise parfois nos marchés. Eh oui ! Je rencontrerai, à l'issue de cette séance au la ministre espagnole de l'agriculture lors d'un « comité mixte franco-espagnol ». Cet espace de concertation nous permettra, je le souhaite, de construire des positions communes pour préserver nos marchés et le fruit du travail de nos viticulteurs. La parole

Un nouveau et énième calendrier de paiement des aides de la PAC a été annoncé par le gouvernement Philippe I en juin dernier, la veille du départ de votre prédécesseur, monsieur le ministre.

Je ne sous-estime pas les raisons qui ont conduit à ces retards, mais j'entends corriger cette situation en prenant des engagements précis et en confinant ce que M. Mézard avait annoncé. Cet engagement est important, parce qu'il s'agit de restaurer le crédit de la parole de l'État auprès des agriculteurs. C'est d'autant plus important que personne, ici et ailleurs, ne méconnaît les difficultés auxquelles sont confrontées, du fait de la baisse des prix à la production, l'ensemble des filières.

J'ai demandé à l'ASP de renforcer sans délai les moyens humains mobilisés pour le chantier de l'instrumentation des aides PAC pour que l'ASP et son prestataire informatique accroissent leur capacité à traiter en parallèle les chantiers du paiement des aides du premier et du deuxième pilier Je veillerai aussi à ce que les services d'économie agricole aient les moyens nécessaires pour traiter ces chantiers en parallèle cet automne.

repris. La campagne de télédéclaration s'étant achevée le 31 mai 2017, il faut réaliser l'instruction des aides 2017 du premier pilier pour permettre leur paiement trésorerie remboursable sera mise en place à la mi-octobre 2017 pour « compenser » le non-paiement des avances et des acomptes versés habituellement en septembre et en octobre. Quant aux campagnes 2018 et suivantes, le calendrier « habituel » sera retrouvé aussi

Certaines estimations faisaient état de plusieurs dizaines de milliers d'hectares de vignes touchés, dont des pans entiers du vignoble du département de l'Aude. Je souhaite donc attirer votre attention sur la situation de détresse des viticulteurs. Certains

toute la mesure de cette catastrophe économique et sociale en mettant en oeuvre en urgence un certain nombre de mesures conjoncturelles et structurelles. Sont attendues

des aides spécifiques exceptionnelles, susceptibles d'être modulées pour les exploitants disposant d'une assurance récolte : il s'agit en fait de permettre aux sinistrés, notamment à ceux d'entre eux qui ne seraient pas assurés, de faire face à leurs besoins immédiats

Par ailleurs, en raison des pertes de marchés qui pourraient s'ensuivre, il est demandé que soient prises toutes dispositions permettant d'autoriser des achats de vendanges par les vignerons sinistrés.

d'une assurance récolte contre les risques climatiques, incluant la grêle ou le gel. Ce soutien prend la forme d'une prise en charge partielle des primes, pouvant aller jusqu'à 65 %.

disponibilité de vins d'entrée de gamme en France. Cette situation suscite des tensions fortes avec nos partenaires et amis Espagnols. Je condamnerai toujours les exactions perpétrées à la frontière franco-espagnole à l'encontre de transporteurs de vins espagnols. Le renforcement en 2016 des enquêtes et contrôles menés par les services des douanes et de la répression des fraudes a révélé la portée limitée des fraudes relevant d'opérateurs français, et l'absence de fraudes de la part des opérateurs espagnols. Malgré cela, ces contrôles se poursuivront en 2017 et en 2018, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché. Enfin, pour

En effet, l'AEFE a décidé de mettre fin à la mise à disposition de logements de fonction dans les locaux adjacents à l'établissement, pour se mettre en conformité avec la loi locale.

selon les délégués du personnel. Pour autant, cette décision de l'AEFE peut entraîner de grandes difficultés pour les personnels du lycée Louis-Massignon, notamment à l'occasion du renouvellement de leur visa. un contrat de location officiel est nécessaire pour l'obtenir. Or il n'est pas rare que les autorités locales expulsent des familles vivant dans des villas partagées

Or, pour des raisons financières évidentes, certaines villas sont aménagées en plusieurs appartements, occupés par différentes familles. Une autre règle applicable à Abu Dhabi est le paiement par avance d'une année entière de loyer, lequel est très élevé.

les autorités françaises ne manqueront pas d'appeler l'attention des autorités émiraties sur l'intérêt qui s'attache à ce que l'établissement puisse continuer à fonctionner avec du personnel de qualité.

ce lycée a un bel avenir devant lui. Des travaux sont prévus pour construire une nouvelle école maternelle, agrandir les espaces extérieurs et rénover les anciens bâtiments.

Ma question porte sur l'état du déploiement des réseaux numériques dans notre pays, sur lequel il convient de faire un point en ce début de quinquennat. Le classement de la France au vingt-septième rang des pays européens pour le très haut débit par la Commission européenne témoigne du retard considérable que nous avons pris.

En matière de déploiement des réseaux mobiles, les objectifs fixés par la loi dite « Macron » n'ont pas été tenus. Selon les derniers chiffres, plus de 550 centres-bourgs attendent encore d'être couverts en 2G,

Le recours à davantage de technologies alternatives à la fibre n'est-il pas un marché de dupes en termes de débit ? Que faut-il penser des annonces de SFR, qui dit vouloir déployer le très haut débit sur l'ensemble du territoire sans argent public ?

C'est comme cela qu'il faut comprendre l'annonce qu'il a faite la semaine dernière devant la Conférence nationale des territoires. Garantir le haut et le très haut débit à tous les Français dès 2020, c'est en réalité poser un jalon intermédiaire

Dans les zones les plus enclavées, là où le déploiement de la fibre est extrêmement coûteux, nous n'aurons d'autre choix que d'utiliser d'autres technologies, au moins pendant une certaine période : le satellite, la boucle locale radio, la 4G fixe.

les objectifs fixés par le Président de la République. SFR a été le premier à répondre, par voie de presse, en promettant de déployer la fibre sur tout le territoire sans argent public.

de « simplifier drastiquement les structures » du Grand Paris et de réunir une conférence territoriale pour aboutir à « une organisation institutionnelle stabilisée et efficace ». Le Président de la République reconnaît ainsi que la création de la métropole sur le périmètre de la petite couronne n'a apporté ni la stabilité ni l'efficacité recherchées.

ici ou là l'idée saugrenue de fusionner les trois départements de petite couronne pour préparer leur « évaporation » au sein de la métropole du Grand Paris. Une telle perspective n'a aucun sens

quels sont donc les projets du Gouvernement pour la métropole du Grand Paris et la place des départements de la petite couronne ? Quelle sera la méthode de concertation ? Quel est votre calendrier ? Monsieur le ministre, la nouvelle majorité a été élue sur la promesse d'un changement des pratiques politiques et sur un engagement de transparence. C'est pourquoi j'aimerais obtenir aujourd'hui l'engagement clair qu'aucune décision ne sera prise sans concertation approfondie et sans l'accord majoritaire des habitants et des élus locaux.

par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, à être regroupés en un seul. Le regroupement est rendu possible par les lois de réforme des collectivités territoriales de 2010 et NOTRe de 2015. Je ne rappellerai pas les débats auxquels j'ai longuement participé : vous connaissez ma position sur la nécessité de maintenir l'échelon départemental, sous

Ces deux départements voisins avaient déjà enclenché, en janvier 2016, un rapprochement, avec la création d'un établissement public interdépartemental, la mutualisation de plusieurs services et la création d'une société d'aménagement. Les objectifs affichés en 2016 par les départements étaient de rationaliser les dépenses de fonctionnement. les dépenses de fonctionnement. Le département des Hauts-de-Seine est inclus dans la métropole du Grand Paris. Celui des Yvelines est membre de l'association Grande Couronne capitale, rassemblant tous les départements de la grande couronne. de la grande couronne. Je précise que la fusion des deux départements ne saurait préempter les choix à venir concernant la métropole du Grand Paris. Ce sujet sera abordé lors de la Conférence territoriale du Grand Paris Paris annoncée par le Président de la République le 17 juillet dernier et qui se tiendra cet automne. D'ici là, nous allons mener une concertation approfondie. Elle est déjà en cours, puisque j'ai commencé

M. le ministre de la cohésion des territoires. La réglementation applicable à ce jour aux autorisations de construire déposées par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les CUMA, est symptomatique des carcans et des freins administratifs que doit supporter le monde agricole. Créatrices de liens de solidarité, les CUMA sont un outil de développement durable de notre agriculture que l'on doit soutenir quand elles envisagent de construire ou d'agrandir des bâtiments nécessaires au stockage ou à l'entretien de matériel. Malheureusement, la jurisprudence a longtemps considéré les CUMA comme des entreprises de services non directement utiles à l'activité économique agricole. Pour cette raison, les CUMA ne pouvaient construire dans les zones agricoles et naturelles des communes. Un exploitant agricole peut le faire, des exploitants agricoles regroupés au sein d'une CUMA n'y sont pas autorisés : cela peut paraître quelque peu paradoxal Nous pensions que la récente recodification du code de l'urbanisme aurait enfin permis de clore ce dossier et de laisser les CUMA réaliser leurs projets. Elle autorise, il est vrai, l'accueil des bâtiments des CUMA dans les zones agricoles et naturelles des communes, mais sous réserve

Au-delà, c'est surtout le sort réservé aux communes actuellement dépourvues de document d'urbanisme ou disposant seulement d'une carte communale qui interpelle. Dans mon département, les Deux-Sèvres, sur un peu plus de 300 communes, un tiers n'ont aucun document d'urbanisme et une soixantaine ne disposent que d'une carte communale. Dans les faits, malgré l'engagement pris par le ministre de l'agriculture de l'époque, la récente recodification du code de l'urbanisme ne permet toujours pas aux CUMA de construire dans les secteurs agricoles et naturels de nombreuses communes soumises au règlement national de l'urbanisme. la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », comporte une disposition qui intéresse le droit de l'urbanisme. Elle vise à faciliter la réhabilitation et l'extension mesurée d'habitations agricoles. Sa rédaction est simple et l'intention qui la

Un travail de réflexion avec la Fédération nationale des CUMA a été conduit par le précédent gouvernement pour faciliter la mutualisation des équipements

28 décembre 2015, qui autorise, dans les zones A et N des PLU, les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériels agricoles par les CUMA. Cette solution d'équilibre permet d'autoriser les constructions et installations des CUMA dont l'implantation en zone A ou N apparaît justifiée, tout en excluant celles destinées à être implantées en zone urbaine, comme les bureaux des salariés des CUMA. Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un PLU, l'implantation de constructions dans les secteurs agricoles et naturels est est également possible. Dans les communes couvertes par une carte communale, il convient de délimiter un secteur constructible destiné à accueillir ces constructions et installations. Quant aux communes communes encore soumises au règlement national d'urbanisme, ces constructions et installations devront faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal, ce qui n'est pas une condition très difficile L'avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers garantira, en outre, l'association des acteurs du monde agricole au choix du secteur d'implantation. En résumé, je vous confirme donc la possibilité, confirme donc la possibilité, dans le cadre établi par le droit actuel, pour les CUMA de construire dans les secteurs agricoles et naturels, y compris dans

des zones de revitalisation rurale, les ZRR, à la suite du décret pris le 16 mars 2017 par le précédent gouvernement, qui a établi une nouvelle liste de communes éligibles à un dispositif largement remanié

intercommunal, et non plus à l'échelle communale, ainsi que deux critères sélectifs, à savoir la densité de population et le revenu par habitant. Ainsi, un grand nombre de communes jusqu'alors intégrées au dispositif sont désormais exclues

ce sursis n'aidera en rien les élus de ces communes à conserver les acteurs et les opérateurs économiques sur leur territoire. Créées en 1995, les ZRR sont un élément fondamental du maillage territorial dans nos départements. droit à un certain nombre d'avantages fiscaux, des exonérations d'impôts nationaux et locaux qui ont jusqu'à présent fait l'unanimité.

à mes services une expertise juridique afin d'examiner les possibilités de limiter les conséquences de la sortie du dispositif. Je travaille sur ce dossier

sont encore trop mal desservis. Or, monsieur le ministre, garantir un accès équitable de l'ensemble des Français aux télécommunications est indispensable à la cohésion entre les territoires vous êtes sensible à cette question. L'État doit donc agir avec les opérateurs pour permettre un déploiement qui tienne compte des spécificités locales.

blanches » ou « grises », qui ne sont couvertes que par un seul opérateur, avec pour conséquence une couverture partielle, voire très partielle, des communes concernées. Dans le département de l'Ardèche, ces problèmes affectent particulièrement les communes de Saint-Laurent-les-Bains, de Laval-d'Aurelle,

dû aux manquements des opérateurs, mais également aux pouvoirs publics, qui tardent à faire construire des pylônes mutualisés permettant l'installation d'antennes relais. L'État a lancé, le 12 décembre 2016, la plateforme France Mobile, opérée par l'Agence du numérique, en y associant les collectivités et leurs élus pour procéder dans les meilleurs délais à l'éradication des zones « blanches » et « grises

Il nous appartient désormais de veiller à ce que les 541 centres-bourgs nouvellement identifiés en zone « blanche » depuis 2016 soient rapidement équipés de nouveaux pylônes qui permettent le déploiement effectif, par les opérateurs, des services mobiles de troisième génération aux habitants. Pour ce faire, l'État a a déjà affecté près de 30 millions d'euros au soutien aux collectivités territoriales. Par ailleurs, nous travaillons à déterminer les modalités d'un meilleur accompagnement de ces collectivités,

avec les collectivités territoriales et les opérateurs de téléphonie mobile. Nous devrons avoir conclu ces travaux avant la fin de l'année, afin d'engager dans les meilleurs délais le plan d'accélération massive

J'ai coécrit un rapport sur ce sujet il y a trois ans, et je parcours la France à l'appel d'élus départementaux désorientés, de responsables de structures aux aguets, de salariés à bout.

explosion des burn-out et des arrêts maladie en lien avec la robotisation des tâches et la perte de sens d'un métier d'abord relationnel. Alors que les salaires sont au plus bas, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement annonçait une revalorisation,

pas totalement appliquées : certains départements retiennent les fonds, d'autres disent ne pas avoir reçu d'enveloppe budgétaire de l'État pour les frais kilométriques, des associations rechignent

Le secteur de l'aide à domicile fait l'objet d'un important soutien de l'État depuis de nombreuses années. L'allocation personnalisée d'autonomie à domicile a été réformée afin de favoriser le soutien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie. À cet égard, vous évoquez des contributions financières nouvelles qui seraient imposées aux bénéficiaires de l'APA. Pourtant, la réforme a permis d'exonérer de participation financière les bénéficiaires les plus modestes, d'alléger le reste à charge des bénéficiaires, en particulier de ceux dont les plans d'aide sont les plus lourds. Elle a revalorisé les plafonds nationaux de l'APA, jusqu'à hauteur de 400 euros par mois pour le niveau de perte d'autonomie le plus élevé. Ces mesures permettent d'augmenter le temps d'accompagnement à domicile et d'élargir la palette de services mobilisables. de leur financement, il est garanti, de façon durable et évolutive, par la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, la CASA. Cette recette nouvelle permet d'accroître la part de la solidarité nationale dans le financement global de l'APA.

Ce fonds d'appui est doté de 50 millions d'euros. Ces crédits peuvent soutenir les départements dans la définition d'une stratégie territoriale d'organisation et de pilotage de l'offre d'aide à domicile, afin de mieux répondre aux besoins.

à domicile, les SAAD, des autres départements peuvent également solliciter l'aide à la restructuration auprès des agences régionales de santé. J'ai annoncé la mise en place d'un groupe de travail qui sera chargé de déterminer le meilleur modèle de financement pour les pour les usagers, en limitant le reste à charge, et d'apporter une réponse pérenne aux difficultés économiques des structures. Ces travaux débuteront dès le mois de septembre. Au-delà des outils mis en place pour accompagner les départements, je poursuivrai le dialogue avec les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. La parole

comptez-vous mettre en oeuvre pour permettre aux structures d'appliquer la loi et de la santé. Madame la ministre, le 8 février dernier, le Conseil d'État a demandé à Mme Marisol Touraine, alors ministre de la santé, de prendre des mesures ou de saisir les autorités compétentes afin d'assurer la disponibilité de vaccins correspondant aux seules vaccinations obligatoires-antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique -prévues aux articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique. La licence d'office est l'une des pistes qu'il a ouvertes en vue de la mise en oeuvre de cette injonction. Le 15 juin dernier, dans une interview au, vous annonciez réfléchir à étendre l'obligation vaccinale à onze valences. Aujourd'hui, madame la ministre, vous semblez avoir fait votre choix. C'est une façon de répondre à la décision du Conseil d'État, mais en la détournant de son objectif premier, me semble-t-il. Alors que la vaccination est une question de santé publique, une protection individuelle et collective indispensable, votre décision inquiète nos concitoyennes et nos concitoyens. concitoyens. La couverture vaccinale est, hélas, en baisse en France, et il est important d'en appréhender les causes, qui sont multifactorielles. Les scandales sanitaires, les liens et conflits d'intérêts mis en lumière, le refus de remise sur le marché de vaccins sans adjuvants aluminiques y sont pour beaucoup. Or votre décision, au lieu de contrer l'obstination des laboratoires à ne pas respecter l'obligation vaccinale en sortant un vaccin à trois valences, valide, dans les faits, leur stratégie. C'est grave, car ces grands laboratoires sont aujourd'hui en mesure d'influencer la politique vaccinale en France, y compris en organisant des pénuries. Madame la ministre, ma question est simple : par quels moyens allez-vous mettre l'industrie pharmaceutique au service de la santé publique, loin des intérêts financiers, et comment allez-vous créer les conditions de la mise en oeuvre de la licence d'office, au moins concernant la production des vaccins ? La parole

L'enjeu est que les Français retrouvent confiance dans la vaccination. La licence d'office n'est pas une solution. Il faudrait qu'un laboratoire ait envie de racheter cette licence d'office et d'investir dans la production d'un vaccin qui n'existerait que pour la France, aucun autre pays ne connaissant d'obligation vaccinale limitée au

ce qu'ont dit les jurys de citoyens et de professionnels de santé lors de la concertation menée par le professeur Fischer : « Les effets indésirables pouvant découler de la vaccination représentent la plus grande crainte liée à la vaccination. Parmi ceux-ci on peut relever les craintes liées aux effets indésirables des sels

au cours des débats sur la loi de modernisation de notre système de santé, un amendement visant à modifier l'article L. 1418-1 du code de la santé publique. Cet amendement tendait à créer, entre l'Agence de la biomédecine et les établissements de santé où sont réalisées les greffes,

Cet amendement devait également permettre d'assurer, s'agissant de la phase sensible des transports, le respect de la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation. Le ministre m'avait répondu qu'un groupe de travail avait été mis en place pour réfléchir à une organisation plus efficiente du prélèvement d'organes dans notre pays et de l'acheminement des greffons

En effet, les systèmes de transport aérien de province et de l'AP-HP ne sont pas coordonnés ; la fermeture nocturne de nombreux aéroports complexifie la manoeuvre logistique ; les militaires, habitués à une chaîne opérationnelle unique et cohérente, se démobilisent ; les hôpitaux exposent des coûts inutiles, qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros ; la sécurité sociale ne bénéficie pas pleinement du moindre coût de la greffe, alors que des dizaines de millions d'euros d'économies sont possibles la solidarité nationale exprimée par les donneurs est gaspillée. Madame la ministre, lors de votre audition devant la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale du mercredi 19 juillet dernier, vous avez fait la déclaration une ministre qui légifère mais qui expérimente. » L'action que je souhaite vous voir entreprendre dans ce domaine correspond parfaitement au nouvel esprit de pragmatisme et d'efficacité qui guide l'action publique. Ma question est la suivante : pouvons-nous simplifier cette procédure en envisageant le plus rapidement possible l'organisation d'une réunion avec tous les acteurs concernés, afin de définir une stratégie pilotée par vous, madame la ministre, d'énoncer la démarche à suivre pour l'Agence de la biomédecine et de les transcrire de manière opérationnelle l'UniHA

vous soulignez à juste titre que le transport d'organes est un des maillons essentiels de notre politique nationale de greffes et qu'il est nécessaire de l'optimiser et de le rationaliser, afin d'économiser des greffons aujourd'hui perdus.

en mars 2017 a permis de définir plusieurs hypothèses d'évolution du modèle de l'organisation des transports. Quatre possibilités ont ainsi été identifiées : mutualiser les moyens des établissements de santé pour les transports, dans le cadre de l'organisation actuelle ; élargir le rôle de l'Agence de la biomédecine

sur les conséquences graves, pour les établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes, de la réforme de la tarification en cours. La situation des personnes âgées dépendantes est, dans notre pays, préoccupante. ans après la création de la journée de solidarité, le service public destiné aux personnes âgées est en danger. En effet, la réforme de la tarification des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes, les EHPAD, actuellement mise en oeuvre, fragilise ce secteur et risque d'avoir un fort impact sur les personnes âgées les plus fragiles et les ménages les plus modestes. Avec plus de 200 millions d'euros de retraits de financement, les établissements publics font face à une situation inextricable qui pourrait, à terme, se traduire par une augmentation du reste à charge pour les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale, au travers d'une libéralisation des tarifs d'hébergement des établissements publics des des déshabilitations ou déconventionnements visant à leur permettre de trouver un équilibre financier. Le contexte de crise a fragilisé les plus exposés, au premier rang desquels se trouvent les personnes âgées et les ménages aux revenus modestes. La réforme en cours vient directement affecter leur quotidien dans un moment de vulnérabilité aiguë. Je demande donc que les modalités de calcul du point des groupes iso-ressources soient réexaminées, et je voudrais savoir quel modèle de financement pourrait être proposé afin d'apporter une réponse globale à la hauteur des enjeux majeurs auxquels il faut faire face. Madame la ministre, je vous remercie de nous faire connaître les intentions précises du Gouvernement sur cette question particulièrement importante pour les personnes âgées accueillies en EHPAD public, leurs familles et les personnels de ces structures, et, plus largement, sur celle de la prise en charge de la dépendance.

un état de dépendance bien plus avancée qu'il y a quelques années. Cela alourdit la prise en charge et amène à s'interroger sur notre modèle de financement. L'objectif de la réforme de la tarification des EHPAD est de rétablir de l'équité dans la répartition des financements au regard des seuls critères de l'état de dépendance et des soins des soins à apporter aux résidants. La réforme organise une convergence progressive des dotations versées par l'assurance maladie au titre des soins et par les conseils départementaux au titre de la dépendance. Afin de ne pas alourdir la charge financière pour les conseils départementaux, la convergence des tarifs « dépendance » des EHPAD est organisée autour du tarif moyen départemental.

crédits doivent accompagner la médicalisation des EHPAD, mais également renforcer la qualité de la prise en charge. Monsieur Milon, j'entends vos inquiétudes. J'ai demandé au directeur général de la cohésion sociale, M. Jean-Philippe Vinquant, de présider un comité de suivi

Faut-il d'autres types de structures ? C'est la question que je me pose. Sur ce point, les travaux engagés par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui doivent être finalisés très prochainement, serviront de base à ma réflexion, en vue de l'élaboration de propositions concrètes. La parole est à M. Alain Milon.

établissement privé à but non lucratif de secteur 1, l'hôpital Marie-Lannelongue, du Plessis-Robinson, bénéficie d'une réputation internationale d'excellence. Son histoire est jalonnée de grandes premières médicales, depuis la greffe coeur-poumons réalisée en 1985 par le professeur Philippe Dartevelle. Cet établissement est aujourd'hui spécialisé dans la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l'enfant et de l'adulte, le traitement chirurgical ou angioplastique de l'hypertension artérielle pulmonaire et la chirurgie des cancers du thorax. Sur ce dernier point, il faut signaler l'étroit partenariat noué avec l'Institut Gustave-Roussy. Grâce à ce partenariat, les patients ont accès aux thérapies et techniques chirurgicales les plus avancées.

Or cette tradition d'excellence a deux conséquences : un taux de recours extrêmement élevé de 37 %, quand la moyenne des centres hospitalo-universitaires est inférieure à 10 un différentiel de coûts de l'ordre de 12,3 millions d'euros, que ni la tarification à l'activité ni la dotation budgétaire au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation ne permettent de couvrir. Malgré une amélioration constante des processus de production et de gestion, l'équilibre financier de l'établissement n'est pas atteint. Dans ces conditions, ma question sera simple, madame la ministre : vous paraît-il envisageable de prévoir un dispositif spécifique et pérenne de compensation permettant à l'hôpital Marie-Lannelongue de faire face aux surcoûts inhérents à l'excellence des soins qu'il assure et de poursuivre l'intégralité de ses activités de recherche ? La parole

Cette diminution de l'activité est liée au départ du chef de pôle, qui a conduit à une perte de recettes de près de 10 millions d'euros en deux ans et à un décrochage

d'activités de recours exceptionnel et à une diminution des financements liés aux publications de l'établissement. La baisse des dotations MERRI avait été compensée intégralement en 2014 par une aide exceptionnelle de l'ARS. Pour autant, l'ARS et le niveau régional n'ont pas vocation à compenser durablement des baisses de financement, qu'elles soient liées au départ d'un chef de pôle ou à une diminution des dotations MERRI.

Ce plan devrait être prêt pour la période de financement 2017-2021 et s'appuyer sur un nouveau projet médical induisant un repositionnement de l'activité de l'établissement et une évolution favorable du. Je le rappelle, plus les établissements sont monothématiques, plus ils sont sensibles à des variations à la baisse des tarifs.

de repenser l'organisation territoriale en faisant reposer cette réorganisation et le plan de retour à l'équilibre sur un projet médical écrit par l'établissement, en vue d'assurer une hausse des recettes d'activités et une meilleure maîtrise des charges. Madame

Ceux qui, par une négligence coupable, n'auront pas permis d'éviter ce drame doivent être jugés et condamnés. Or, aujourd'hui, pour une vingtaine de dossiers déposés avec le soutien de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, les conclusions récentes de l'instruction ouvrent la voie vers un non-lieu, et donc vers une absence de procès. Les juges estiment qu'il est impossible de dater le moment de la commission de la faute, et donc d'imputer celle-ci à quiconque. Cette décision est particulièrement grave pour les victimes de l'amiante, qui sont en droit d'attendre réparation mais aussi transparence absolue sur les négligences constatées. Les industriels qui ont sciemment prolongé l'utilisation d'un matériau qu'ils savaient mortel, ceux qui ont laissé faire et les lobbyistes du comité permanent amiante, qui ont milité contre l'interdiction, doivent être jugés. Il est arrivé que des décisions et des orientations aient été prises par des décideurs économiques en pleine conscience des dégâts humains et environnementaux qu'elles impliquaient. En conséquence, ces crimes industriels doivent être impérativement instruits et jugés en tenant compte de la gravité des fautes commises. Toutes les leçons de cette catastrophe doivent être tirées afin que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent jamais plus de telles tragédies. Car, au-delà de la question de l'amiante, cela pourrait signifier que pour d'autres produits que l'on emploie aujourd'hui dans l'industrie, ou encore pour les pesticides, par exemple, nous serions susceptibles d'avoir les mêmes décisions juridiques dans vingt ou trente ans. Ce n'est pas possible ! Madame la ministre, notre démocratie, vous le savez, traverse une période de grande fragilité. C'est pourquoi les prises de position sur un sujet aussi sensible sont attendues avec impatience et une forme d'espérance. Partant du principe que les pollueurs par l'amiante, comme les pollueurs par tout autre produit dangereux, devraient être les payeurs, je souhaite savoir, madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet sensible de santé publique.

Vous interrogez le Gouvernent sur les cancers liés à l'amiante. Comme vous le rappelez, la justice a été saisie, et il ne m'appartient pas de commenter ses décisions. Il est très important d'indemniser les victimes pour le préjudice qu'elles ont subi. C'est la raison pour laquelle le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, a été créé voilà plus de quinze

des actions concertées entre les administrations impliquées. Les travaux s'organisent autour de cinq axes : renforcer et adapter l'information des professionnels ; améliorer et accélérer la professionnalisation ; faciliter et accompagner la mise en oeuvre de la réglementation liée à l'amiante ; soutenir et promouvoir les démarches de recherche et de développement sur l'amiante se doter d'outils de connaissance, de suivi et d'évaluation. Depuis peu, un site interministériel dédié à l'amiante est accessible sur le portail du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Il est également possible de consulter le bilan de la mise en oeuvre des actions de ce plan interministériel

les règles d'évaluation des risques et de mise sur le marché sont définies dans un cadre réglementaire européen. Il convient de vérifier que la liste des produits à risque est régulièrement mise à jour

Je tiens à vous assurer que l'État prendra toutes ses responsabilités et édictera les mesures nécessaires pour éliminer progressivement l'utilisation des pesticides dans l'environnement. Sachez également que, dans ma stratégie nationale de santé, qui vise à promouvoir la prévention, les questions de

Madame la ministre, le patrimoine immobilier de nos villes et de nos petites cités de caractère nécessite une attention toute particulière afin qu'il puisse être conservé pour les générations à venir. Il existe, à cette fin, plusieurs dispositifs permettant de donner aux propriétaires privés les moyens de réaliser des travaux de sauvegarde ou de restauration. compte cependant d'un cas particulier : celui des villes à secteur sauvegardé, qui ne peuvent disposer des aides de la Fondation du patrimoine, au prétexte qu'elles bénéficient de la loi Malraux. Or cette loi ne garantit plus les avantages fiscaux prévus initialement à destination des propriétaires occupants.

visait à simplifier et à moderniser la protection de notre patrimoine. Elle n'a malheureusement pas apporté de solution à ce problème particulier des villes à secteur sauvegardé. Dans certaines communes, les bâtiments qui auraient besoin d'être restaurés sont occupés par leurs propriétaires, qui sont donc privés de tout soutien financier. Les biens se dégradent rapidement. C'est une partie importante du patrimoine qui est menacée. Ma question, madame la ministre, est la suivante : le Gouvernement est-il favorable à l'élargissement du dispositif d'aide de la Fondation du patrimoine aux sites patrimoniaux remarquables- c'est la nouvelle dénomination des villes à secteur sauvegardé -, afin de permettre aux propriétaires occupants de pouvoir financer équitablement les travaux auxquels ils sont soumis ? Quelles sont, de manière générale, les mesures concernant la préservation du patrimoine qui sont envisagées

vous m'interrogez sur l'éligibilité aux aides de la Fondation du patrimoine des villes à secteur sauvegardé. Comme vous le savez, le ministère de la culture, tout comme le Parlement, est particulièrement attentif à la protection et à la mise en valeur des ensembles urbains et paysagers C'est pourquoi, par souci de clarification et d'efficacité, la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite « loi LCAP », a regroupé sous l'appellation de « sites patrimoniaux remarquables » les anciens « secteurs sauvegardés les anciennes « aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine », et les anciennes « zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager À la suite de cette évolution des outils de protection du patrimoine, et dans ce même objectif de simplification, nous avons souhaité, en lien avec Bercy, mettre en cohérence les dispositifs fiscaux associés de deux manières. Dès la loi de finances rectificative pour 2016, nous avons permis d'appliquer à ces sites patrimoniaux remarquables la fiscalité dite « Malraux », en vigueur dans les anciens dispositifs. La seconde mesure- c'est l'objet de votre question, monsieur le sénateur -consiste en une révision de la doctrine fiscale en faveur du patrimoine. En effet, j'ai le plaisir de vous annoncer ce matin que l'ensemble de ces nouveaux sites patrimoniaux remarquables seront désormais éligibles au label délivré par la Fondation du patrimoine aux propriétaires privés pour des travaux, ainsi qu'aux déductions fiscales au titre de ces travaux.

Enfin, vous me permettrez, j'en suis sûre, de profiter de cette question pour saluer dans cet hémicycle le travail remarquable de la Fondation du patrimoine qui, grâce à son implantation territoriale, à l'action de ses bénévoles et à ses interventions sur le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, conduit une action exemplaire,

actuellement bloquées. Dans ses premières semaines à la tête du Gouvernement, le Premier ministre a indiqué qu'il considérait comme « élevé » le coût de tels contrats, et qu'il souhaitait, dès lors, ne continuer d'y recourir que « de façon maîtrisée ». Les emplois d'avenir ont été créés en 2012 ; ils ont pour objectif de faciliter l'insertion sur le marché du travail des jeunes peu ou non qualifiés en leur proposant un emploi à temps plein de longue durée incluant un projet de formation. Le bilan établi à la fin de l'année 2016 prévoyait que, un an après la signature de leur contrat, trois jeunes en emploi d'avenir sur quatre auraient bénéficié d'une formation, et qu'un sur deux aurait certifiante. Cet accès plus facile à la certification résulte d'un effort de formation qui bénéficie notamment aux non-diplômés et aux plus jeunes. Ainsi, plus de 325 000 contrats d'emplois d'avenir ont été signés depuis 2012 et 51 % des jeunes

dialogue social. Madame la sénatrice, vous interrogez le Gouvernement au sujet des emplois d'avenir. Le soutien à l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés du marché du travail, notamment des jeunes, est une priorité du Gouvernement, priorité qui doit toutefois tenir compte de l'amélioration de la conjoncture économique ainsi que de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Vous le savez, les emplois d'avenir visent à lutter contre la précarité professionnelle des jeunes peu ou non qualifiés, en rupture avec le monde éducatif. Leur mobilisation doit donc s'articuler avec la palette d'outils que le Gouvernement entend conforter afin que chaque jeune trouve la réponse à son besoin, à son projet. Ainsi, en matière de formation, les jeunes seront l'un des publics prioritaires du plan d'investissement dans les compétences. Nous souhaitons également renforcer, faciliter et sécuriser l'accès à l'apprentissage et la réussite de ces parcours en développant les dispositifs permettant d'amener les jeunes en difficulté vers l'alternance, puis de les accompagner, pour éviter les ruptures de contrat. En matière d'accompagnement intensif, la garantie jeunes portée par les missions locales et l'accompagnement intensif des jeunes vont enfin poursuivre leur montée en puissance. Dans ce cadre, le volume d'emplois d'avenir a donc vocation à diminuer. Pour l'année 2017, le volume total de contrats s'élèvera à plus de 39 000, soit 4 000 contrats de plus que ne le prévoyait la loi de finances initiale.

l'opportunité de transposer certains paramètres des emplois d'avenir aux autres catégories de contrats aidés. Enfin, nous souhaitons renforcer une approche décloisonnée de l'ensemble de ces outils, qui doit servir la logique de parcours du jeune. La parole

Plusieurs maires de communes nouvelles ont fait savoir qu'ils rencontraient des difficultés du fait de l'absence de prise en compte de la réduction de la part départementale de la taxe d'habitation, ce que l'on au moment des votes des taux de fiscalité de la commune. Or la loi ne prévoit aucun dispositif particulier pour empêcher le risque de hausse de la taxe d'habitation pour les ménages.

Les services de la direction générale des collectivités locales comme ceux de la direction générale des finances publiques ont identifié ce problème, qu'ils qualifient d'anomalie, et ont proposé une solution les communes nouvelles concernées qui souhaitent corriger leur politique fiscale votée en 2017 sont invitées à prendre rapidement contact avec les services préfectoraux ou avec les services de la direction départementale des finances publiques. Ils reçoivent alors un nouvel état 1259 comprenant le débasage du taux de taxe d'habitation. Elles bénéficient d'un délai supplémentaire pour délibérer leurs taux de fiscalité pour 2017. Un nouveau vote peut effectivement intervenir, mais, dans ce cas, les recettes de la commune sont amputées à due concurrence de la baisse des taux votée par le conseil municipal.

ministre, je souhaiterais du moins que vous puissiez apporter aux communes nouvelles concernées par cette anomalie toute garantie que la solution fiscale proposée cette année est claire et sécurisée. de l'intérieur. Monsieur le sénateur Michel Vaspart, vous appelez mon attention sur l'augmentation de la taxe d'habitation à l'occasion de la création de communes nouvelles et notamment sur la situation de la commune nouvelle de Beaussais-sur-Mer dans votre département, les Côtes-d'Armor. Bien qu'il soit effectivement lié au transfert de la part départementale de la taxe d'habitation au bloc communal lors de la réforme de la taxe professionnelle intervenue en 2011, le sujet que vous évoquez ne relève pas d'une problématique de taux, mais se rapporte aux abattements. Le transfert de la part départementale de la taxe d'habitation a en effet donné lieu à la correction, à la hausse ou à la baisse, des abattements communaux et intercommunaux, afin qu'ils intègrent ceux qui étaient en vigueur au sein de la part départementale à la date de la réforme. Cela est évidemment obligatoire. Or, en cas de création d'une commune nouvelle- c'est le cas que vous soulevez -, les abattements de taxe d'habitation applicables sur le territoire des anciennes communes sont soit harmonisés sur délibération de la commune nouvelle,

Il en résulte qu'une commune nouvelle peut voir la taxe d'habitation augmenter sur son territoire, faute de délibération pour harmoniser son régime d'abattement ou parce que le nouveau régime d'abattement a été harmonisé sans tenir compte des corrections d'abattement. Pour corriger cet effet, la commune nouvelle de Beaussais-sur-Mer aurait pu harmoniser ses abattements en prévoyant, comme le permet l'article 1411 du code général des impôts, de majorer d'un ou de plusieurs points l'abattement pour charge de famille, puisque c'est de cela qu'il s'agit. En tout état de cause, le conseil municipal peut délibérer avant le 1 octobre 2017 pour augmenter les abattements applicables sur son territoire à compter de 2018.

Madame la ministre, mon interpellation de ce matin s'inscrit au coeur d'une actualité criante dans l'ensemble du territoire départemental, du Chablais à la frontière genevoise, de la vallée de l'Arve aux bords du lac d'Annecy ou dans l'Albanais. d'ailleurs bien volontiers mes collègues Jean-Claude Carle et Cyril Pellevat, présents tous les deux ce matin pour entendre votre réponse. Sur le terrain, les habitants, les entreprises et les agriculteurs subissent les effets des installations illicites quand les forces de l'ordre et les élus ne sont plus en mesure de maîtriser la situation. Celle-ci révèle notre incapacité collective à agir, elle décrédibilise l'action de l'État et celle de la justice, tout cela alors que ce phénomène prend une ampleur considérable, partout et de manière récurrente. Les élus locaux ont mis en place, en investissement qu'en fonctionnement, des aires d'accueil pour les petits et les grands passages. Même si ces obligations sont issues de la loi et du schéma départemental, ils ont eu besoin d'un grand courage politique pour faire passer de telles décisions- je parle ici en connaissance de cause, et président d'intercommunalité. À l'heure où je vous parle, il me semble pertinent de revisiter la loi Besson, de requalifier certaines incriminations pénales et de simplifier les procédures administratives et judiciaires. Madame la ministre, nous sommes en plein été et la Haute-Savoie connaît une activité touristique importante, l'un des piliers de notre économie dans cette région frontalière et de montagne. Quelles initiatives le Gouvernement compte-t-il prendre en la matière dans les mois qui viennent ? Quel travail pouvons-nous construire ensemble, en nous fondant sur la proposition de loi déposée par notre collègue Jean-Claude Carle ou sur celle que je vais déposer cette semaine ? Par ailleurs, au moment où la Haute-Savoie connaît une situation aussi critique, quels moyens pourraient être alloués par le ministère de l'intérieur pour y remédier ? La parole

vous m'alertez sur la situation problématique des occupations illicites de terrains par les gens du voyage en Haute-Savoie, cet été. L'installation d'un certain nombre de groupes au comportement irrespectueux sur des terrains agricoles ou sur des zones industrielles, situés parfois à proximité des zones d'habitation, suscite évidemment des tensions avec la population.

Ces installations illicites entretiennent la confusion, voire l'amalgame, entre ces groupes et la majorité des gens du voyage, qui s'installent sur les aires d'accueil dédiées et ne provoquent pas de troubles. Bien sûr, quand les gens du voyage respectent la loi, il faut

Dans le même temps, il faut pouvoir effectivement lutter contre les occupations illicites. En Haute-Savoie, les demandes d'expulsion à la suite d'une occupation illicite ont augmenté de 50 % depuis un an. Les outils juridiques disponibles doivent être utilisés au maximum, et je demande aux préfets d'agir en ce sens : vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle toutefois que l'évacuation des occupants illicites est conditionnée, pour la commune demandeuse, au fait d'avoir satisfait à ses obligations au titre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage- c'est tout à fait le

à la citoyenneté a ainsi abrogé tout titre de circulation, un progrès demandé depuis longtemps, et a prévu une adaptation des obligations des collectivités locales pour tenir compte de la sédentarisation

qui devront être apportées cette année. Toutefois, soyons bien clairs, si les objectifs du schéma départemental sont atteints dans l'essentiel du territoire de la Haute-Savoie, jamais notre département ne pourra accueillir tous les groupes de voyageurs qui voudraient s'y installer.

en ma qualité de rapporteur spécial du budget de la mission « Justice » pour la Haute Assemblée, je ne connais que trop vos problématiques budgétaires, mais je souhaite appeler votre attention sur le nécessaire maintien d'une présence judiciaire équilibrée sur nos territoires, en particulier dans le département de l'Aisne, que je représente ici. modernisation de la justice du XXI siècle, les ministères de la justice et des affaires sociales ont rendu conjointement, en février 2016, un rapport sur le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TASS, des tribunaux du contentieux de l'incapacité, ou TCI, et des commissions départementales d'aide sociale,

Or, bien que soulignant, d'une part, que le département de l'Aisne compte deux TASS, l'un à Laon, l'autre à Saint-Quentin, et que, d'autre part, la comparaison des affaires en stock entre ces deux juridictions montre une meilleure évacuation des affaires au tribunal de Laon, ce rapport prévoit prévoit pourtant l'absorption du TASS de Laon par celui de Saint-Quentin. Cette disposition aboutirait à la concentration exceptionnelle d'un pôle économique et social dans cette ville au détriment de la ville préfecture, ainsi fi de l'éloignement géographique qui augmenterait considérablement pour de nombreux justiciables- parfois plus de 200 kilomètres aller-retour -, de l'efficacité avérée du TASS de Laon, et des locaux du conseil de prud'hommes de Laon, qui ont la capacité logistique et immobilière d'accueillir le TASS de Laon au sein d'un pôle cohérent et efficace.

le rapport interministériel que vous évoquez énumère effectivement le cas de départements dans lesquels existent actuellement plusieurs tribunaux de grande instance et où le contentieux social

au sein d'un pôle social constitué dans un TGI par département. Néanmoins, à ce stade, je tiens à vous le dire, monsieur le sénateur, aucune décision n'est prise quant à l'implantation des futurs pôles sociaux.

des TCI, des cours d'appel, des CDAS, des caisses primaires d'assurance maladie, des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale. Ces comités ont notamment un rôle d'analyse de la situation de chacune des entités concernées et ont fait remonter à la Chancellerie, ces dernières semaines, leurs observations. La désignation des juridictions qui assumeront le rôle de pôle social s'appuiera bien entendu sur les conclusions de ces comités locaux, qui sont en cours d'analyse par mes services

Je peux néanmoins vous assurer que je veillerai au maintien de l'équilibre judiciaire territorial dans votre département et que je serai extrêmement attentive à la proximité et à l'accessibilité des différentes juridictions.

puisque, pour des contentieux qui relèvent actuellement du TCI d'Amiens, ils pourront à l'avenir se rendre au pôle social du TGI de leur département. Il me semble donc que, de ce point de vue, il y aura une amélioration de l'accessibilité. La parole

était dans les années 1960 la plus rapide de France, souffre d'équipements devenus vétustes et de retards chroniques. En outre, il est quasiment impossible d'y utiliser les réseaux internet et de

C'est pourquoi je souhaiterais obtenir un certain nombre de précisions quant à la modernisation des matériels roulants. Quel est l'état des travaux à ce jour ? Où en est l'appel d'offres européen concernant les futures rames ? Quand celles-ci seront-elles livrées ? J'insiste tout particulièrement sur le fait que, à la suite de l'abandon du projet de création de la ligne Paris-Poitiers-Limoges, la ligne POLT constitue désormais l'unique axe ferroviaire entre l'ancienne région Limousin et Paris. Elle revêt donc une importance considérable en matière de désenclavement géographique et donc d'avenir économique des départements, le plus souvent ruraux, qu'elle dessert. Aujourd'hui, l'arrêt du lancement de lignes à grande vitesse redonne toute leur place à ces lignes traditionnelles, comme celle du POLT,

sera rendu public et si un certain nombre de mesures préconisées seront retenues dans l'élaboration de la future stratégie. Enfin, les élus locaux se demandent si les lignes transversales vont être conservées,

et aux malades hospitalisés au CHU de cette ville. Cette question des lignes subsidiaires n'est pas anecdotique, dans la mesure où 60 % des voyageurs utilisant le POLT en sont issus. Les membres de la représentation nationale concernés par tous les territoires situés entre Brive, Limoges et Paris,

pour améliorer le confort et la qualité de service qui y sont proposés. Ainsi, 500 millions d'euros seront consacrés à la modernisation de son infrastructure sur la période 2015-2020, ce qui représente un doublement par rapport au rythme d'investissement de la période 2005-2014. À cet important effort de régénération, dont le rythme sera maintenu sur la période 2020-2025, viendront s'ajouter plus de 120 millions d'euros d'investissements inscrits dans les contrats de plan État-régions 2015-2020, pour améliorer la fiabilité et la régularité des temps de parcours. Par ailleurs, comme vous le savez, un appel à candidatures en vue d'acquérir un matériel au confort adapté aux parcours de moyenne et longue distances a été lancé à la demande de l'État par SNCF Mobilités en décembre dernier. L'appel d'offres est en cours et la procédure se poursuit. Cette amélioration du confort des voyageurs est particulièrement nécessaire sur cet axe structurant

je diffuserai très prochainement le rapport de M. Delebarre et je vous proposerai une réunion à la rentrée, avec les collectivités concernées, pour que nous puissions examiner ensemble les pistes définies dans ce rapport.

L'ensemble de ces éléments va permettre d'alimenter le schéma directeur de la ligne pour proposer des mesures visant à améliorer le service de cet axe. Je peux vous assurer que le Gouvernement est mobilisé sur les transports du quotidien, d'assurer une mobilité pour tous dans tous les territoires et permettre à chacun de bénéficier d'une mobilité alternative à la voiture. Toute cette démarche s'inscrit pleinement en cohérence avec les orientations présentées par le Président de la République, notamment la priorité accordée à l'entretien et la régénération des réseaux existants.

Situés le long de la Seine, les ports du Havre, de Rouen et de Paris sont reliés directement à l'arc atlantique et constituent donc de formidables portes d'entrée pour le commerce extérieur français. Or les ports de l'axe Seine, réunis au sein du GIE HAROPA, sont en concurrence directe avec les ports du nord de l'Europe, Rotterdam, Anvers et Hambourg. Plusieurs facteurs handicapent aujourd'hui les ports normands et, plus globalement, les ports français. Ces handicaps tiennent notamment à la gouvernance, aux règles d'occupation du domaine public maritime, à la fiscalité, aux aides de l'État ou encore aux infrastructures. La qualité des infrastructures est une condition indispensable pour étendre l'portuaire. L'exemple du port d'Anvers, deuxième port d'Europe, qui poursuit et amplifie ses investissements dans les infrastructures fluviales et ferroviaires, témoigne de la nécessité de s'adapter pour capter toujours plus de marchés. Tout y est mis en oeuvre pour favoriser l'attractivité du port, qui voit l'activité de son nouveau terminal à conteneurs monter en charge.

En comparaison, le port du Havre achemine 80 % de ses marchandises par la route, 15 % par le transport fluvial et 5 % seulement par le fret ferroviaire. Or la concentration des acteurs maritimes et le gigantisme des navires entraînent une mutation forte du transport maritime, qui impose aujourd'hui une véritable massification des moyens de transport des conteneurs. La densification par le transport ferroviaire, moins coûteux et plus respectueux de l'environnement, est essentielle pour maintenir la compétitivité des ports français, d'autant que la loi relative à la transition énergétique la programmation pluriannuelle de l'énergie, ont mis l'accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment celles de CO2. Le report du transport de marchandises de la route vers le fret ferroviaire est aujourd'hui essentiel ; il s'inscrit dans cette démarche. Les enjeux justifient l'évolution de nos infrastructures ferroviaires pour mieux connecter les ports de l'axe Seine à l'européen. De plus, la compétitivité des ports nécessite aujourd'hui l'élaboration d'une véritable politique maritime et portuaire qui valorise les atouts maritimes. Madame la ministre, j'aimerais savoir quelles seront vos premières décisions pour montrer cette volonté de renforcer la compétitivité des ports normands et donner à notre pays une véritable politique maritime portuaire.

Le renforcement de la compétitivité de nos ports est un enjeu stratégique fort. Vous pouvez compter sur moi pour m'atteler, dans les mois qui viennent, à leur développement. Comme vous l'avez évoqué, cela passe par un ensemble de mesures.

se coordonnent pour former un acteur portuaire intégré, attractif et durable. Il faudra également refonder le modèle économique de nos ports pour leur donner les moyens réels de leur développement. je serai notamment attentive à la clarification des relations financières et fiscales entre l'État et ses établissements publics portuaires.

européens. Comme vous l'avez souligné, il faut aussi soutenir la desserte massifiée de nos places portuaires. Au sein du port du Havre, l'État, en investissant aux côtés du port et des collectivités pour la construction d'un nouveau terminal multimodal, a soutenu un véritable outil industriel, industriel, même s'il faut encore développer le trafic et enrichir les services offerts par ce terminal. Ainsi que vous l'avez indiqué, la compétitivité d'un port dépend également de sa capacité à desservir son arrière-pays par les transports terrestres. il est vrai que le mode ferroviaire n'occupe pas la place qu'il devrait avoir dans la desserte du port du Havre. Cette situation doit évoluer dans les prochaines années et le Gouvernement y est pleinement engagé. Ainsi, les premiers travaux de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors-Pontoise viennent de débuter. Il s'agit de créer un itinéraire fret alternatif à celui de l'axe historique de la vallée de la Seine, actuellement proche de la saturation. La mise en service est attendue à l'été 2020.

ligne cumule un manque d'entretien et bien d'autres handicaps, tels que la présence de 111 passages à niveau sur 168 kilomètres et trop peu de zones d'évitement. Pourtant, Pourtant, elle constitue l'un des axes ferroviaires majeurs du département, avec 700 000 usagers annuels. L'état actuel de l'infrastructure ne permet plus

En 2013, une estimation réalisée par SNCF Réseau chiffrait le montant des travaux à réaliser à 45 millions d'euros. La première tranche de ces travaux avait même été inscrite dans le contrat de plan État-région 2015-2020, actant une participation aux deux tiers par l'État et la région et, pour le tiers restant, par les collectivités locales concernées et SNCF Réseau. Mais, le 20 juin dernier, une nouvelle étude commandée par l'entreprise ferroviaire voyait bondir le coût de cette réhabilitation à 91 millions d'euros, rebattant les cartes de la répartition précédemment envisagée. Ainsi, à l'inquiétude et à la frustration des usagers, largement laissés pour compte dans ce dossier, vient s'ajouter le désarroi des élus, qui l'ont manifesté lors de l'inauguration de la LGV Bordeaux-Paris, en attendant de vous, madame la ministre, des garanties quant à la réalisation et au financement de ce projet par l'État. L'arrivée de la LGV à Bordeaux et Libourne devait constituer, entre autres, une formidable opportunité pour nos concitoyens périgourdins : celle de bénéficier de temps de trajets réduits vers la capitale. Or force est de constater que ni l'état de l'infrastructure ni le cadencement des trains ne le permettent

s'inscrit pleinement dans le souhait du Gouvernement d'accorder la priorité à l'entretien et à la régénération des lignes existantes et aux transports de la vie quotidienne. Comme vous l'avez rappelé, des études ont été réalisées, préalablement au contrat de plan État-région, sur la possibilité d'améliorer la desserte de Bergerac et son raccordement au réseau à grande vitesse Libourne et Bordeaux. Les travaux de régénération de cette ligne sont inscrits au contrat de plan État-région 2015-2020, selon une clé de répartition que vous avez mentionnée. Ils devront permettre d'assurer la pérennité de l'infrastructure entre Libourne et Bergerac et donc d'éviter la mise en place de ralentissements, qui seraient très pénalisants pour les voyageurs. que vous le soulignez, la dernière estimation de l'opération s'élève à environ 91 millions d'euros, montant que le maître d'ouvrage explique par une dégradation accélérée de l'état de la plateforme ferroviaire. Des optimisations du programme et des coûts sont certainement encore possibles. Elles seront étudiées dans le cadre d'un groupe de travail spécifique.

Néanmoins, l'État est prêt à réaffecter les crédits selon les priorités qui seront définies par la région. Il faudra donc que le préfet de région examine avec les représentants des collectivités territoriales les possibilités de parvenir à un nouveau plan de financement, dans le respect des principes que je viens d'évoquer. En outre, maintenant que l'opération Sud-Europe-Atlantique est terminée, SNCF Réseau va pouvoir réaffecter des ressources humaines en fonction des priorités définies par la région sur les actions de sécurisation et de fiabilisation du réseau.

D'ailleurs, une douzaine d'associations se sont prononcées contre ce projet et, lors des réunions d'information, les populations concernées ont exprimé leur refus

représentant 70 000 habitants directement touchés par ce tracé de contournement et farouchement opposés à sa mise en oeuvre. Les motifs d'opposition sont divers et fondés. De fait, il paraît inconcevable de faire l'impasse sur les questions d'environnement,

Il porte également atteinte à l'économie et à l'emploi, en menaçant de détruire, s'il est mené à son terme, une zone foncière de 400 hectares, ainsi qu'une zone d'activité économique où sont employés plusieurs centaines de salariés.

au Conseil d'État. La commission d'enquête a rendu un avis favorable sur le projet, en soulignant qu'il répondait à des objectifs qui lui avaient été fixés, notamment par sa capacité à délester l'hypercentre de Rouen. En réponse à certaines de ses réserves et recommandations, des mesures complémentaires ont été intégrées au projet, en particulier en matière de qualité de l'air, de maîtrise des nuisances sonores et d'insertion dans l'environnement. S'agissant des modalités de financement du projet, elles ont été partagées avec les collectivités territoriales concernées. Elles sont, du reste, exposées dans le cadre du dossier de l'enquête publique. Il est ainsi envisagé que ce projet, estimé à 886 millions d'euros, soit réalisé sous le mode concessif, avec une mise à péage. Néanmoins, une subvention publique d'équilibre, estimée à 55 % du coût est nécessaire, les recettes de péage ne permettant pas de couvrir l'ensemble des coûts de construction de cette infrastructure. À ce stade, ce projet est concerné, comme l'ensemble des grandes infrastructures hors contrat de plan État-région, par la « pause » annoncée par le Président de la République le 1 juillet dernier. Comme nous l'avons déjà évoqué dans cette assemblée, l'addition des engagements pris par les précédents gouvernements conduit, en effet, à une impasse de 10 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. Les Assises de la mobilité que je lancerai en septembre viseront à identifier les besoins de chaque territoire, à examiner les ressources mobilisables, en répondant à un impératif : celui d'adapter les besoins et les ressources. Elles permettront de préparer le projet de loi d'orientation sur les mobilités, qui sera présenté au Parlement 2018 et qui comprendra à la fois une vision à moyen terme des infrastructures et une programmation quinquennale des investissements, équilibrée en ressources et en dépenses et prenant mieux en compte la priorité à l'entretien et à la maintenance des réseaux existants.

chenilles processionnaires urticantes, des punaises de lit ou encore des rats, les nuisibles envahissent de plus en plus espaces verts, exploitations agricoles, forêts, villes et villages, logements, le risque qu'en soient importés davantage des quatre coins du monde étant accru durant la période des vacances d'été.

Dans nos communes, les particuliers se tournent très naturellement vers leur maire, souvent désemparé face à un fléau qui ne connaît pas de frontières et qui peut conduire à l'hospitalisation des personnes touchées et à des chocs allergiques chez les animaux. À cela s'ajoute la restriction- totalement justifiée -d'utilisation des solutions biocides pour raisons environnementales, mais qui rend les traitements moins efficaces. Et les essais menés sur les territoires n'en sont encore qu'à un stade expérimental.

on estime à 38 millions d'euros par an les coûts engendrés par les nuisibles en France. Madame la secrétaire d'État, face à un fléau qui appelle la mise en place urgente de moyens de lutte à la fois techniques et financiers à l'échelle nationale

Vous venez d'évoquer plusieurs espèces dont la prolifération a des conséquences directes non seulement sur la faune sauvage et domestique, mais aussi sur l'homme. Depuis plusieurs années, l'État met en place des mesures de régulation adaptées. Je pense, par exemple, au frelon Arrivé accidentellement en France en 2004, il s'est largement installé sur le territoire national et a rapidement montré son caractère invasif et dommageable, notamment vis-à-vis des abeilles domestiques. La loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété le code de l'environnement pour agir efficacement contre ce type d'espèces exotiques envahissantes. Le décret publié le 23 avril 2017 a permis de préciser les dispositions de contrôle et de gestion de leur propagation. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le frelon asiatique a été classé en danger sanitaire de catégorie 2 et que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation finance des études pour évaluer les moyens de faire baisser la pression de prédation. Vous avez également évoqué le moustique tigre, espèce invasive installée en France depuis 2004 et qui peut être vecteur de maladies telles que la dengue et le chikungunya.

La politique préconisée pour lutter contre la chenille processionnaire s'appuie sur une gestion localisée et ciblée impliquant une responsabilisation des pouvoirs locaux et des particuliers.